monsieur le président.

aux bailleurs, consentis dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, en les assimilant à des subventions d'équilibre ou de fonctionnement non soumises à la TVA. Les subventions et aides financières aux bailleurs viennent compenser tout ou partie des pertes de loyers et peuvent être accompagnées de conditions relatives au maintien d'une activité économique, culturelle ou associative locale souvent fragile. En l'état actuel du droit, ces soutiens financiers risquent d'être assimilés à des modalités de paiement des loyers par un tiers au locataire et soumis de ce fait à la TVA. Il est observé que la base d'imposition correspondant à ces aides n'entraînera pas de TVA déductible chez le locataire, produisant de fait un gain fiscal pour l'État financé par les collectivités territoriales. Il est ainsi proposé de corriger cet effet d'aubaine non anticipé et de sécuriser juridiquement l'aide des collectivités aux bailleurs afin qu'ils consentent aux abandons de loyers encouragés par l'État.

l'avis du Gouvernement ? Au-delà de la pertinence de l'amendement, le cadre juridique de l'Union européenne n'autorise pas les États membres à modifier les éléments à comprendre dans la base d'imposition à la TVA, tels qu'ils sont décrits à l'article 73 de la directive TVA. Cette assiette inclut notamment les subventions, qui sont la contrepartie de la livraison d'un bien ou d'une prestation de service rendue au profit de la partie versante. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cette considération. Au demeurant, la qualification d'une somme comme subvention complément de prix taxable est une question qui ne s'apprécie qu'au cas par cas et en fonction des circonstances de l'espèce. Pour ce faire, les conditions d'une telle qualification sont strictes : le principe du versement de la subvention doit exister en droit ou en fait avant l'intervention du fait générateur des opérations dont elle constitue la contrepartie, et le prix du bien ou du service doit être déterminé, partant de ce principe, au plus tard au moment où intervient le fait générateur de ces opérations.

est extrêmement coûteuse en trésorerie. Il nous paraît plus opportun de cibler nos efforts sur des plans sectoriels de relance de l'activité. Au-delà, votre proposition consiste à étendre les effets du système d'amortissement dégressif, qui est une exception au principe général d'amortissement linéaire fondé sur les annuités d'amortissement de montant constant, et nous considérons que ce dispositif n'a pas vocation à être élargi de manière aussi générale. Nous craignons même que le dispositif que vous proposez puisse créer un effet d'aubaine important, notamment pour des entreprises des secteurs les moins touchés

Le Gouvernement affiche des objectifs ambitieux en matière écologique, notamment sur les véhicules.

jusqu'au 31 décembre 2020 le mécanisme de suramortissement dont bénéficient les entreprises pour l'acquisition de véhicules propres. La promotion de la transition énergétique passe par l'essor de formes de mobilité moins émissives et moins polluantes il s'agit d'un enjeu de premier ordre puisque le secteur des transports concentre à lui seul 29,9 % de nos émissions de gaz à effet de serre, le précédent budget carbone ayant par ailleurs été dépassé de 8,1 % dans ce secteur. Pour y parvenir, la demande privée doit être mobilisée à plein, ce qui suppose d'aider les entreprises à constituer des « flottes captives » de véhicules propres. Or, le plan de soutien à la filière automobile se contente essentiellement d'élargir, pour les ménages, les critères d'éligibilité à la prime à la conversion.

étendu la dépense fiscale liée au dispositif de suramortissement en faveur des véhicules lourds sur plusieurs points, et le dispositif a été prorogé de deux ans jusqu'en décembre 2021 ; le taux de suramortissement a été porté à 60 % pour les véhicules dont le poids est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, et il a été étendu à un certain nombre de véhicules. Le Gouvernement est attaché à cet équilibre. Il nous semble que les dispositions votées pour 2019 et pour 2020 rendent ce secteur suffisamment attractif. C'est la raison pour laquelle l'avis est défavorable.

suite de la crise du covid. Par ailleurs, la délégation sénatoriale aux entreprises avait déjà réalisé un travail sur le sujet. Son rapport sur l'utilisation du numérique dans les PME PME avait mis en exergue un défaut dans ces structures par manque à la fois de moyens et de formation. Cet amendement vise à répondre à ces deux problématiques en instituant pour cinq ans

à Mme Jacky Deromedi. Cet amendement crée un crédit d'impôt pour lequel les entreprises industrielles pourront opter si elles ne choisissent pas le suramortissement. Il s'agit d'une initiative bienvenue, qui résulte des auditions menées conjointement pendant le confinement par la commission des affaires économiques et la délégation aux entreprises. En outre, ce crédit d'impôt est ouvert à toutes les PME,

de celles des professionnels du secteur, qui ont mis en évidence le rôle essentiel que devront jouer les robots d'assistance physique pour les PME artisanales dans les prochaines années. Il s'appliquerait également aux formations liées à l'acquisition d'un équipement numérique, conformément à une autre recommandation du rapport d'information sur l'accompagnement de la numérisation des PME et TPE, et à la proposition de l'Autorité des normes comptables (ANC), de décembre 2019, de modifier le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, afin de rendre une partie de la formation amortissable. Enfin, il prendrait en compte l'abonnement à des logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation, le mécanisme actuel ne concernant que l'acquisition de ces logiciels. Les entreprises recourent de plus en plus à ce modèle d'exploitation commerciale, commerciale, le, dans lequel les logiciels sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Les clients ne paient pas de licence d'utilisation pour une version, mais utilisent librement le service en ligne ou, plus généralement, paient un abonnement. Ces motifs conduiront le Sénat, je n'en doute pas, à adopter des mesures propres à conforter les investissements des PME, lesquels sont cruciaux pour amplifier la relance de notre économie.

au nombre desquels il faut citer la déduction prévue par l'article 39 B du code général des impôts, mais vous avez pris la peine de préciser que les deux dispositifs ne sont pas cumulables, ou le crédit d'impôt formation des dirigeants. J'ajoute que les PME soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé au nombre desquels les logiciels, les machines de production à commande programmable ou numérique, ou encore les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation. Le champ est donc extrêmement large. L'article 244 M du code général des impôts prévoit aussi un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite de 40 heures de formation par année, et les actions de formation s'étendent notamment de l'adaptation et du développement des compétences à l'acquisition, à l'entretien et au perfectionnement de ces compétences. Par ailleurs, onze opérateurs de compétences agréés sont chargés d'accompagner la formation professionnelle et de financer l'apprentissage ; ils aident les branches à construire leur certification professionnelle en la matière.

dépassant la règle de la durée maximale de quatre ans. Je partage en cela la prudence exprimée par le rapporteur général sur la création de nouveaux crédits d'impôt. Enfin, dernier point que je veux soulever pour solliciter le retrait des amendements le fait que le texte prévoie un renvoi à un décret pour préciser les catégories de prestations et d'équipements éligibles nous paraît comporter un risque d'incompétence négative qui serait sanctionné par le Conseil constitutionnel. Donc, pour

La faible dynamique observée aujourd'hui en matière de cession-transmission découle d'une politique de soutien aux entreprises trop orientée vers les créations d'entreprises. Il importe de procéder à un rééquilibrage des avantages, en particulier fiscaux, vers la reprise d'entreprise. le plan fiscal, il importe d'adopter deux mesures incitatives pour doper la reprise des PME et ETI industrielles, si importante pour le devenir de nos territoires, si chers à notre Premier ministre. La première mesure consiste à créer un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d'entreprises visant notamment les PME. Une seconde mesure consister à réévaluer le plafond d'exonération de l'impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d'une petite ou moyenne entreprise appartenant à une branche d'activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. S'agissant de la majoration du plafond d'exonération, le surcoût devrait être de 25 millions d'euros. Ainsi, on peut raisonnablement estimer que le coût du présent amendement serait de 81 millions d'euros par an. Dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous connaissons actuellement, il est urgent d'adopter un tel dispositif. J'ajoute que cet amendement met en oeuvre l'une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti socialiste et ses deux groupes parlementaires.

du Gouvernement ? C'est un peu la même problématique que celle des véhicules poids lourds. L'amendement de M. le rapporteur général conduira à remettre en cause des dispositions adoptées l'an dernier visant à une conformité avec le droit communautaire. Il nous semble que cet amendement conduirait à une remise en cause de la conformité, compte tenu de l'intensité de l'aide, supérieure à celle prévue par la réglementation des aides d'État, puisque nous serions à 42 %, avec une déduction de 150 %, compte tenu d'un taux d'IS à 28 Or le plafond communautaire est fixé à 40 % des coûts éligibles. Donc au-delà de notre attachement aux équilibres trouvés l'an dernier, nous craignons que cela aille au-delà des règles communautaires. Par ailleurs, nous considérons aussi que cette mesure

Cuypers. Cet amendement a pour objet d'instituer une déduction fiscale de 40 % sur l'impôt sur les sociétés (IS) et l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour l'utilisation des biocarburants aéronautiques par les compagnies aériennes. L'effort consenti en direction des biocarburants aéronautiques est encore déclamatoire. Certes, plusieurs initiatives récentes sont à saluer, comme la conclusion d'un engagement pour la croissance verte relatif à la mise en place d'une filière de biocarburants aéronautiques durables en France. Pour autant, le Gouvernement n'a pas encore déployé de moyens à la hauteur de ces enjeux. Or le secteur du transport aérien représente un débouché de premier ordre pour les biocarburants. Ceux-ci constituent une solution précieuse pour décarboner les avions,

Par ailleurs, leurs gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre s'élèvent à 90 % par rapport au kérosène classique. Pour autant, des freins à l'essor des biocarburants aéronautiques subsistent toujours.

vise à instituer une déduction fiscale de 40 % sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'acquisition et l'installation d'infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburants alternatifs qui sont ouvertes au public. Or les mesures prévues dans ce domaine par le plan de soutien à la filière automobile concernent exclusivement les bornes de recharge électriques ouvertes au public, avec un objectif de déploiement de 100 000 bornes d'ici à 2021, en particulier autour des grands axes nationaux. Dans ce contexte, il est impératif d'aller plus loin pour développer la mixité des véhicules propres en favorisant l'ensemble des carburants alternatifs et de garantir la couverture de tout le territoire

(LOM) a instauré au bénéfice des salariés du secteur privé effectuant tout ou partie de leur trajet domicile-travail à vélo, en covoiturage ou en transports en commun. La prime est facultative pour l'employeur et plafonnée à 400 euros par an.

et d'autoriser le cumul entre l'exonération de charges au titre du remboursement des transports en commun et au titre du forfait mobilités durables. Notre amendement tend à reprendre ces propositions. La parole

monsieur le ministre, que l'on peut attendre un peu puisqu'un projet de loi est prévu à l'automne. Mais certaines mesures pourraient opportunément être mises en oeuvre dès maintenant. Ce serait un bon signal.

Mettez-vous à leur place : s'ils utilisent la voiture, c'est parce que les transports en commun ou le vélo sont moins pratiques. En plein mois de juillet,

ou du temps ! Soyons raisonnables, et faisons confiance à nos concitoyens ! À l'État d'organiser correctement les transports en Île-de-France pour que chacun

Lurel. Les membres du groupe socialiste et républicain demandent au Sénat de mettre fin à une injustice infligée à Saint-Martin

tous les départements d'outre-mer bénéficient d'un taux d'aide fiscale à l'investissement de 53,55 %, sauf Saint-Martin, dont le taux s'élève à 45,9 %. À l'époque, monsieur le ministre, à la même place, vous aviez expliqué que Saint-Martin n'en avait pas besoin

et d'adopter cet amendement.

issue du mécénat en 2020 aura des conséquences dramatiques sur le financement de l'ensemble des lieux et structures de diffusion culturelle et de création artistique et sur l'entretien et la conservation du patrimoine. Le nouveau régime fiscal issu de la loi de finances pour 2020, créant un plafond de 2 millions d'euros, au-delà duquel le mécénat d'entreprise pouvait être défiscalisé à 40 %, au lieu de 60 % précédemment, risquait déjà de réduire les ressources financières à disposition des différents secteurs artistiques, culturels et patrimoniaux. Face à la crise liée au covid-19, il convient de de recalibrer les outils fiscaux permettant de participer au financement de la culture et du patrimoine. Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à relever le taux de défiscalisation des dépenses de mécénat à hauteur 60 % pour l'année 2020. Cela permettra de gommer les effets

De fait, ils ont souvent perdu l'activité qui leur permettait de maintenir leurs ressources et ne peuvent bénéficier d'aucune aide par ailleurs. Leur seul recours est donc l'appel aux dons. Dans ce contexte, il serait opportun de permettre une réduction d'impôt plus importante pour les dons effectués au profit de ces organismes afin de leur permettre de pérenniser leurs actions d'intérêt général. L'amendement

Non seulement ils ne bénéficient pas d'un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique, mais ils ne rentrent dans aucun dispositif d'aide proposé par le Gouvernement, notamment notamment les producteurs fermiers. Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d'être écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire, et que certains circuits de vente n'ont pas encore été Afin de soutenir les dons et d'indemniser le mieux possible les pertes considérables des producteurs, le présent amendement crée un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l'exercice du premier semestre 2020. Ce dispositif temporaire permettra ainsi de soulager utilement ces filières professionnelles, qui se sont justement organisées pour garantir l'excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Il s'agit de protéger un fleuron de l'agroalimentaire français. La parole

l'amendement n° 578. Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de denrées alimentaires qui, face au manque de débouchés en raison du confinement, ont multiplié les dons aux organismes caritatifs de leurs productions périssables. Cela est particulièrement vrai pour les fruits et légumes, mais aussi pour les fromages sous AOP et IGP ou pour les fromages fermiers, qui, en raison de la fermeture des rayons de coupe en grands magasins et sur les marchés pendant le confinement, ont été pour partie donnés à ces associations, dans la mesure où 90 % de ces fromages ont une durée de conservation n'excédant pas huit semaines. Afin de soutenir les dons et d'indemniser le mieux possible les pertes importantes des producteurs, le présent amendement vise à créer un dispositif temporaire de défiscalisation renforcée des dons alimentaires sur une grande partie de l'année 2020, au-delà de la période de confinement, notamment pour faire face à l'afflux important de personnes relevant du dispositif de l'aide alimentaire en raison de la crise économique. La

de réduction d'impôt au-delà de 2 millions d'euros. La Cour des comptes, dans un rapport de 2018, a pointé que, en l'espace d'une petite quinzaine d'années, de 2004 à 2017, la dépense fiscale liée au crédit d'impôt mécénat a été multipliée par dix, passant de 90 millions d'euros qu'elle est concentrée à 44 % sur 24 sociétés, et que seules 78 sociétés dépassent les 2 millions d'euros de mécénat par an.

Monsieur le ministre, Or il nous semble que l'abandon de la condition tenant à l'absence de changement significatif de l'activité, notamment en termes d'emploi, et son remplacement par une seule condition d'objectif environnemental ne se justifie pas si le maintien de l'emploi peut être justement concilié avec l'objectif écologique. Aussi, cet allégement de conditions nous paraît assez excessif

Bocquet. Avec cet amendement relatif à la taxation des grands groupes du numérique, nous sommes au coeur de l'actualité. En effet, chacun sait que, cette semaine, le Tribunal de l'Union européenne a

avec cet amendement d'y remédier afin que chacun apporte sa nécessaire contribution au redressement des économies mondiales.

du Gouvernement ? Plusieurs dispositifs déjà en vigueur- je pense notamment à l'ordonnance de report des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire ou encore à la jurisprudence sur la force majeure -permettent de couvrir des situations de retard de chantier quand des délais sont imposés pour des raisons fiscales. Le report de deux ans du délai d'achèvement proposé par les auteurs de cet amendement ne nous paraît pas opportun dans le cadre des dispositifs que nous examinons. Le mécanisme arrivant à échéance à la fin de l'année, il ne s'agit que de couvrir des projets déjà lancés du fait des retards liés à la crise, non pas d'assouplir le dispositif pour de futurs projets. Ce sont les deux raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En conséquence, à court terme, l'urgence doit être de soutenir la trésorerie de ces entreprises. Il serait nécessaire qu'une partie des factures non acquittées par les microentreprises, à l'issue du report de paiement prévu par la loi d'urgence sanitaire, soient prises en charge par l'État au titre de la solidarité nationale.

Bienvenue, cette baisse du taux de l'IS devait permettre de combler partiellement un écart qui s'est creusé avec les pays concurrents, plaçant la France au tout premier rang pour la hauteur des taux. Sa mise en oeuvre, étalée sur plusieurs années, avait semblé hésitante. Mes doutes n'ont pas manqué de se confirmer : compte tenu du coût budgétaire des mesures prises en réaction au mouvement des « gilets jaunes », le Gouvernement a décidé en 2019 de reporter la baisse de l'IS pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions d'euros. Rappelons pourtant qu'avec un taux normal d'IS abaissé à 25 % à l'issue du quinquennat, la France continuerait à avoir un taux supérieur à la moyenne européenne, qui s'établit à 23 %. à 23 %. À situation inchangée dans les autres États membres de l'Union européenne, dix-neuf d'entre eux auront même en 2022 un taux inférieur à 25 %. On a reporté la baisse uniquement sur les grosses entreprises, laissant une fois de plus entendre que les gros pouvaient payer. Mais c'est oublier que l'impôt payé par ces grandes entreprises est toujours supporté au bout du compte par les consommateurs, les salariés ou encore les fournisseurs. Ce sont les lois de l'incidence fiscale : celui qui paie l'impôt n'est pas toujours celui qui en supporte la charge, et c'est particulièrement vrai s'agissant des impôts sur les entreprises. Cet amendement vise ni plus ni moins à en revenir à la trajectoire de baisse initialement prévue. Il tend en quelque sorte à inviter le Gouvernement à respecter son engagement et la parole donnée. Quel

Or le taux effectif constaté en 2014 est de 0,005 % ! Soit 13 milliards de moins dans les caisses de l'Irlande ! Aux États-Unis, l'excellent Donald Trump, en arrivant aux affaires, a fait passer le taux de l'impôt sur les sociétés de 39 % à 15 %. Est-ce votre modèle ?

Je vais être très clair : elle ne sert à rien ! On peut donc gagner 5 milliards d'euros assez facilement ! Je vous y encourage. Et la pédagogie étant l'art de la répétition, nous proposons à nouveau la suppression de la

des déficits, ou, permet à l'entreprise de constater un profit exceptionnel non taxable, d'améliorer son résultat comptable et ses fonds propres et sa trésorerie lors du remboursement. Pour aider les entreprises à faire face à la crise et leur permettre de rebondir au plus vite, il est proposé de permettre l'imputation des déficits des années 2020 et 2021 sur les bénéfices des trois exercices précédents et de porter la limite d'imputation de 1 million à 5 millions d'euros. Par ailleurs, la créance issue de ce dispositif au titre des exercices clos en 2020 bénéficiera des dispositions de remboursement anticipé prévues à l'article 2 du présent projet de loi.

une telle mesure a été évoquée lors des débats à l'Assemblée nationale. Au regard de l'allocation des moyens dont nous disposons pour financer la relance, il nous paraît prématuré de préempter ces 450 millions d'euros en

Pour les oeuvres audiovisuelles, le plafond du crédit d'impôt a été relevé de 1 300 à 3 000 euros par minute pour les oeuvres d'animation et peut atteindre 10 000 euros par minute pour les oeuvres de fiction. De même, le taux du crédit d'impôt a été relevé à 30 % pour les oeuvres cinématographiques d'animation et les oeuvres cinématographiques réalisées principalement ou intégralement en langue française.

Que la crise ne nous fasse pas oublier que, malheureusement, le changement climatique est toujours une lourde menace ! Or l'un des principaux responsables est le dioxyde de carbone, qu'émet, vous le savez, tout déplacement utilisant un moteur thermique.

Cette taxe est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Sa mise en oeuvre s'appuie sur un dispositif normatif qui existe déjà le décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport. Ce texte impose aux transporteurs de fournir le volume d'émissions de chaque opération à leurs clients. Dès lors, cette évolution est plus facile à envisager. Les chargeurs, eux-mêmes informés précisément de leurs émissions de CO2 par leurs prestataires de transport, feront une déclaration directe de leur volume d'émissions de CO2

acceptabilité. Ce principe peut facilement être reproduit pour contribuer à réduire l'impact du transport sur l'environnement. Il aura ensuite la charge de redistribuer les recettes ainsi encaissées à l'ensemble des parties prenantes et de l'État, pour entretenir et rénover les infrastructures de transport nationales et encourager la transition énergétique de tous les modes de transport de marchandises.

ainsi qu'à des actions de sensibilisation et de formation des donneurs d'ordre et des transporteurs. À l'heure de l'urgence écologique et de la relance verte de notre économie, cette contribution envoie un signal net aux donneurs d'ordre : revoir leurs circuits de distribution. Elle incite toute la filière à revoir ses circuits logistiques sans pour autant punir les entreprises de transport, qui ne sont, en définitive, que des intermédiaires dans la chaîne de livraison. Quel

Le Gouvernement le répète à l'envi, il faut plus que jamais prendre en compte l'impératif écologique dans nos choix budgétaires. Avec cet amendement, nous proposons de créer une véritable contribution écologique, selon le principe pollueur-payeur, au service de la transition énergétique et du report modal. ce titre, les entreprises qui décident du transport, les donneurs d'ordre, doivent être redevables d'une éco-contribution visant la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d'orientation des mobilités. Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant, d'un impact limité pour le choix de meilleures solutions plus écoresponsables et tournées vers les énergies propres, cette éco-contribution est une véritable solution pédagogique pour les donneurs d'ordre et pérenne pour le financement, l'entretien et la rénovation des infrastructures. Elle permettra de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l'environnement, qu'il suffit d'appliquer. Elle donne un coût à la tonne de CO2 déclarée aux donneurs d'ordre par les transporteurs. En l'occurrence, pour obtenir la même recette que l'exonération de 2 centimes par litre qui a fait débat à la fin de l'année 2019, il conviendrait de fixer à 6,30 euros le prix d'une tonne de carbone.

de manière progressive, en prévoyant que soient taxées les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu'un point de retrait ou un établissement du fournisseur. Nous prévoyons également de dispenser de cette taxe les livraisons qui se font dans les communes de moins de 20 000 habitants, pour ne pas pénaliser les tissus moins denses, notamment la ruralité. prévoyons de ne pas taxer les jeunes entreprises du commerce qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, moins de dix salariés et un bénéfice inférieur à 60 000 euros. Il s'agirait d'une taxe de 1 euro pour les livraisons de biens n'excédant pas 100 euros, de 2 euros entre 101 et 1 000 euros et de 5 euros pour les biens d'une valeur supérieure à 1 000 euros.

De ce fait, leurs bilans vont être déséquilibrés et leurs ratios de solvabilité vont se dégrader, ce qui peut rendre l'accès au crédit et aux assurances crédit plus difficile et plus cher. Certaines entreprises disposent de plus-values latentes sur leurs actifs immobilisés. Cet amendement a donc pour objet d'autoriser une réévaluation des actifs immobilisés de ces entreprises, avec une neutralité fiscale des plus-values pouvant être constatées.

un crédit d'impôt transitoire jusqu'au 31 décembre 2021 sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d'événements sportifs, afin de les inciter à conserver, voire à accroître, leurs engagements en faveur du sport alors que les clubs sont fortement touchés par la crise. Le sponsoring sportif et ses activations font partie des budgets de communication que la crise actuelle met en danger. Ils constituent entre 20 % et 50 % des revenus des détenteurs de droits et sont indispensables à la survie du secteur. Sans incitation envers les annonceurs, une baisse d'investissements des sponsors de 28,6 % pour la période 2020-2021, semblable à celle subie lors de la crise de 2008, est à redouter, selon une enquête d'impact conduite par Sporsora auprès de ses membres ; et le retour à un rythme normal d'investissements en communication et sponsoring ne pourrait s'opérer avant 2022. Il convient donc de sécuriser les ressources des clubs sportifs professionnels et amateurs, lesquels ont été durement touchés par la crise, et de favoriser la relance de leurs activités.

est l'avis du Gouvernement ? Même avis. La loi de finances pour 2020 a déjà prévu un mécanisme permettant de stabiliser le nombre de logements PLS éligibles au crédit d'impôt, en retenant pour la détermination du quota de 25 le nombre moyen de logements livrés sur une période de trois ans. Cette méthode permet de prévenir les effets d'une variation exceptionnelle des livraisons de logements au titre d'une année particulière, laquelle serait imputable à des circonstances indépendantes du besoin réel. Nous tenons à l'équilibre ainsi trouvé.

les opérations de démolition réalisées en vue de construire de nouveaux logements sociaux.

Si votre demande concerne un étalement purement comptable, elle n'a pas vocation à figurer dans un texte fiscal ; c'est le code de commerce et l'Autorité des normes comptables qui fixent les règles en la matière. En outre, étaler l'aide fiscale n'est pas compatible avec l'objectif d'une mobilisation précoce du montant de ce crédit d'impôt, comme le montre son mécanisme d'imputation et de restitution. Ainsi, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 X du code général des impôts est imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel le fait générateur du crédit d'impôt est survenu. Si son montant excède l'impôt dû, le crédit d'impôt est restitué immédiatement. Par ailleurs, pour des besoins de trésorerie immédiate, les organismes de logement social ont la possibilité de céder ou d'amortir leurs créances futures de crédits d'impôt avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés. Nous ne partageons donc pas l'opportunité de la mesure que vous proposez,

ce montant est bien trop faible pour avoir un effet dissuasif. L'objectif de cette proposition est donc d'augmenter cette éco-contribution afin de mieux refléter les dommages environnementaux générés par l'aviation. La parole

Le scrutin est ouvert.

est à M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à proposer pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de trois par rapport à celle qui est perçue pour les autres véhicules. Cette taxe serait due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Quel

doivent disposer de véhicules 4x4 pour leurs besoins opérationnels : feux de forêt, inondations ou recherches de personnes en milieu accidenté, par exemple. Un véhicule communément utilisé de marque non française, dont le prix d'achat sur le marché est de l'ordre de 35 000 euros, donne ainsi lieu à une dépense de 11 500 euros sur le budget de fonctionnement du SDIS. Le renforcement du malus écologique est évidemment positif, il est urgent de pousser les particuliers à acquérir des véhicules plus propres alors que l'on sait que l'augmentation du poids des véhicules ces dernières années annule complètement les économies d'essence dues aux moteurs.

pour le climat. Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et le poids du véhicule. Afin que le soutien au secteur automobile soit cohérent à la fois avec l'urgence climatique et avec les aspirations des citoyens à la transition écologique, il est nécessaire d'envoyer un signal clair, dès aujourd'hui, aux producteurs et aux consommateurs. En effet, le malus est aujourd'hui trop faiblement dissuasif et ne permet pas de décourager l'achat de véhicules trop émetteurs de CO2. Au total, moins de 5 % des véhicules subissent un malus de plus de 1 000 euros. De plus, la prise en compte des émissions de CO2 n'est pas suffisante pour rendre compte de l'impact environnemental d'un véhicule : comme le souligne le rapport de France Stratégie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelles n'ont quasiment pas baissé

de la transition des flottes de véhicules vers l'électrique. C'est pourquoi il est proposé ici d'intégrer un « malus poids » en supplément du malus lié aux émissions de CO2. Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu'il n'appliquerait de « malus poids » qu'aux véhicules de plus de 1 400 kilos, ou de 1 000 kilos pour les véhicules électriques ou de 1 700 kilos pour les véhicules hybrides, un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s'appliquer qu'aux plus lourds. Enfin, au-delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV ont une dangerosité accrue pour les piétons et les cyclistes, consomment davantage d'espace public au détriment des autres usagers et leur freinage émet davantage de particules fines, ce qui justifie également de décourager leur achat. Je précise, pour finir, que, comme souhaité par la Convention citoyenne, cet amendement prévoit un ajustement du malus pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.

J'espère que les membres de la Convention citoyenne pour le climat nous écoutent. La droite a manifestement décidé de faire litière de leurs propositions

que le Parlement ne soit pas seulement à la remorque de l'initiative gouvernementale, nous ne devrions pas organiser à la rentrée un débat dans cet hémicycle sur le thème : qu'est-ce qui relève de la croissance verte ?

pour connaître les effets de l'oxyde de soufre. Nous avons donc un devoir de précaution : il faut, d'un côté, encourager les études pour essayer de se protéger des effets négatifs et, de l'autre, mettre à contribution ceux qui utilisent

M. le ministre

la même exonération de taxe sur les véhicules de sociétés qu'aux véhicules dont la motorisation fonctionne au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié.

vise en outre à instaurer un seuil de tolérance de cinq jours dans le calcul de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, la TSVR, pour la période du confinement. Comme le prévoit l'article 284 du code des douanes, l'utilisation temporaire des véhicules de plus de 12 tonnes permet de solliciter une régularisation au temps de non-circulation. Ce calcul s'effectue au mois : lorsqu'un véhicule est en circulation une seule journée au cours du mois, la TSVR est due pour le mois complet ... Compte tenu

La communication de cette déclaration est également simplifiée par la diminution du nombre de pièces demandées. Enfin, la déclaration par courriel est possible pour toute l'année 2020, une mesure de simplification qui gagnera à être pérennisée.

à raison. Par ailleurs, dans la mesure où nous avons autorisé la déclaration d'arrêt temporaire des véhicules jusqu'au 30 juin 2020, soit assez au-delà de la période de confinement, les entreprises qui ont vu des véhicules arrêtés ont pu déclarer ces arrêts et bénéficier des dispositions qui accompagnent cette déclaration. J'ajoute

des entrepôts du commerce électronique, c'est-à-dire des surfaces de stockage non attenantes à un commerce physique. Cette mesure concernerait les surfaces de plus de 400 mètres carrés et les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 460 000 euros. Je redoute, évidemment, que le rapporteur général ne réponde qu'il s'agit plutôt d'un débat de projet de loi de finances

confinement. La période de confinement a été extrêmement favorable au commerce électronique, qui s'est massivement développé au détriment du commerce physique.

pour ne pas citer la multinationale Amazon. Ce contexte aggrave la situation de concurrence déloyale dont souffre le commerce de proximité, pourtant essentiel à la vie des territoires, face au commerce en ligne. Dans une situation d'urgence économique et sociale, cet amendement vise, comme les précédents, à rétablir une concurrence plus loyale entre le commerce de proximité et les grandes plateformes de e-commerce, en soumettant les entrepôts logistiques destinés à la vente en ligne qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail à la taxe sur les surfaces commerciales. Il faudra bien qu'on y arrive ! Cet amendement a également pour objet, dans un contexte d'urgence environnementale, de contribuer à lutter contre l'artificialisation des sols. l'annonce récente du Président de la République, reprise par le Premier ministre, d'un moratoire sur les aménagements de zones commerciales périurbaines est pour un certain nombre d'entre nous une excellente nouvelle. Mais les entrepôts d'e-commerce seront-ils également concernés par ce moratoire ? Les propos tenus par le Président de la République restent flous à ce sujet. Il serait pourtant plus que cohérent afin de préserver les sols non artificialisés et les services écosystémiques qu'ils fournissent, mais aussi de prévoir un traitement équitable entre le commerce physique de proximité et le commerce en ligne.

De la même manière, les entrepôts des acteurs du e-commerce qui appartiennent à un groupe dont la présence physique, au travers de ses autres entités, contribue à la fiscalité territoriale ne seraient pas redevables de cet élargissement de la Tascom.

la disposition que vous proposez, qui est identique à une disposition proposée à l'Assemblée nationale, exonère de cette taxe les entrepôts logistiques qui sont adossés à des surfaces de commerce, sans qu'il y ait de critères pour caractériser celles-ci. Il suffirait qu'un des géants que vous voulez cibler

les commerces qui contournent les ventes habituelles. Pendant le confinement, j'ai interpellé un ministre- en visioconférence, bien évidemment -sur la distorsion de concurrence qui était en train de s'installer entre le commerce physique et, notamment, Amazon. Il m'a été répondu

du commerce électronique- je partage en cela les remarques et les réflexions de la présidente Primas sur les différences qu'il convient de faire entre les différents acteurs et leur mode d'intervention -, à ce stade, la disposition proposée ne nous paraît pas

La cession-bail est une opération financière qui permet à une entreprise, quelle que soit sa taille, propriétaire d'un actif immobilier de le vendre à un crédit-bailleur au prix du marché. En contrepartie, le crédit-bailleur lui consent un contrat de location-vente. Pendant la période de location, le vendeur paie un loyer ; à l'issue du contrat de bail, il récupère la propriété de son actif immobilier. Cette opération présente deux avantages. Premièrement, elle permet à une entreprise de ne pas se dessaisir définitivement d'un actif immobilier. C'est le cas, par exemple, du petit hôtelier ou bien du petit restaurateur, qui est attaché à son actif,

traduite dans le passé par une diminution nette de 30 millions d'euros de la part territoriale des subventions de fonctionnement aux clubs et au mouvement sportif amateur dans les territoires et par une diminution de 30 millions d'euros du cofinancement des équipements sportifs. L'amendement vise à répondre à ces demandes de remise à niveau : aides aux clubs et soutien au financement des équipements sportifs. Je crois que l'urgence nous impose de déplafonner ces deux taxes.

qu'il s'agisse du haut niveau ou de la pratique amateur.

Si le choc est conjoncturel, il est aussi révélateur des problèmes structurels qui frappent l'île. L'auteur de l'amendement prévoit une simple mise à jour des bénéficiaires de la compensation des pertes de recettes issues de la TEOM à Mayotte, compensation de la minoration de 60 % de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation à Mayotte. Il s'agit de faire bénéficier les EPCI à fiscalité propre mahorais de cette compensation, puisqu'ils perçoivent la TEOM. La loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer ne les avait pas inclus, car, à l'époque, la TEOM n'était perçue que par un syndicat mixte à Mayotte, d'où l'actualisation proposée.

entre les entreprises propriétaires de leurs machines et celles qui les louent sous la forme d'un crédit-bail, ces dernières pouvant différer leurs charges.

elles aussi, aux conséquences des restrictions de circulation mises en place pour lutter contre l'épidémie de covid-19 : fermeture ou désorganisation des marchés et des circuits de commercialisation. Les acteurs de ces secteurs économiques n'ont pas pu écouler leur production dans des conditions normales et constateront de fait une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de l'exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

que les producteurs de vins et de spiritueux ont subi de plein fouet.

de mauvais augure sur la viticulture, comme la taxe Trump, la chute des marchés internationaux et la fermeture des restaurants à cause de l'épidémie de covid-19, a empêché nombre de producteurs d'écouler leur production. Il y a donc stockage et, quand il y a stockage de la production, il y a imposition sur les stocks de produits invendus. Cet amendement vise à mettre en place, à titre exceptionnel, un dispositif d'atténuation de l'impact fiscal et social de ce « surstockage ». Nous proposons que ce mécanisme puisse être activé sur décision de l'opérateur et ne concerne que l'exercice 2020. Il bénéficierait à toutes les exploitations redevables de l'impôt sur le revenu sur les sociétés. Il s'appliquerait donc au résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais au revenu professionnel servant d'assiette aux cotisations sociales des agriculteurs. Je vous remercie d'accéder à notre demande de soutien à la viticulture française.

est du même avis. Nous avons pris un certain nombre de dispositions pour aider la viticulture, qui ont été complétées à deux reprises.

monsieur le président.

ou la déduction pour épargne de précaution, mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, devraient pouvoir l'utiliser dès maintenant Toutefois, afin que le montant des prélèvements liés à l'utilisation de ces sommes n'ait pas d'impact négatif et n'entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, nous proposons un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences du recours à la fois à l'épargne au titre de la DPA et de la DEP sur le résultat fiscal réalisé en 2020 et sur le revenu professionnel 2020, qui servira d'assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

en des dispositifs de défiscalisation des bénéfices agricoles, ce qui n'est pas acceptable pour des questions juridiques, comme l'a expliqué le rapporteur général. Madame

on l'a dit, un grand nombre de dispositifs fiscaux allant du fonds de solidarité pour les petites entreprises au chômage partiel en passant par les prêts garantis par l'État. Ces dispositifs existent et ont été adoptés, me semble-t-il, à une très large majorité.

amendement. À titre d'exemple, le commerce de gros spécialisé dans l'approvisionnement du bâtiment a perdu plus de 65 % de son chiffre d'affaires, celui de la restauration publique et commerciale 80 % à 90 % de son chiffre d'affaires.

rien d'autre que des complexifications de la procédure existante. Les entreprises agricoles sont déjà contrôlées, sur facture, pour leur usage de carburant, afin de prétendre au remboursement partiel de TICPE. Aussi cet amendement vise-t-il à supprimer toute référence à une liste de machines au gazole ou à un registre de chantiers.

Ces derniers sont actuellement imposés dès l'année de leur perception, sans tenir compte du rythme d'amortissement du bien faisant l'objet de l'investissement. Cette disposition est très pénalisante pour l'entreprise qui investit dans la transition énergétique : elle paie, de fait, un surplus d'impôt. le présent amendement, d'étaler le paiement selon le rythme d'usage du bien. Le dispositif n'implique pas de déperdition fiscale. De plus, il se révèle

l'entrée en vigueur de la suppression du taux réduit de taxe intérieure sur les produits énergétiques sur les carburants « sous condition d'emploi ». Les taxes intérieures de consommation sur l'énergie fossile et la TVA de 20 % sur la fiscalité énergétique s'élèvent à 47,03 milliards d'euros en 2018, soit 2,3 % du PIB. Cela représente un désavantage compétitif pour les entreprises, la France étant classée au premier rang des grands pays européens en termes de taxation implicite de l'énergie. Or, loin du « gel » annoncé dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020, le Gouvernement a augmenté de 3,9 milliards d'euros la fiscalité énergétique, dont 2,4 milliards d'euros pour les ménages et 1,5 milliard d'euros Selon les éléments d'évaluation du projet de loi de finances pour 2020, la suppression du taux réduit de TICPE sur les carburants « sous condition d'emploi » représente ainsi une charge fiscale pour les entreprises de 200 millions d'euros dès 2020 et de 870 millions d'euros à compter de 2023.

Si les biocarburants routiers et aéronautiques font l'objet d'une prise en compte grandissante de la part des pouvoirs publics, il en va différemment de ceux qui sont utilisés pour le chauffage. Afin d'accompagner le verdissement des chaudières au fioul, encore utilisées par quelque 4 millions de foyers, un tarif réduit de TICPE sur le biofioul à usage domestique serait bien utile dans cette période.

dont bénéficient les biocarburants les plus incorporés, en appliquant un taux de 6,43 euros par hectolitre à l'ensemble d'entre eux, soit les B100, les E85 et les ED95. Les filières françaises de biocarburants sont durement affectées par la crise. Les ventes de biocarburants ont chuté parallèlement à celles des carburants fossiles. La France, de même que ses concurrents, a dû constituer des stocks importants de biocarburants. À titre d'exemple, aux États-Unis et au Brésil, les stocks d'éthanol atteignent neuf mois de consommation, avec un prix inférieur d'un quart à la normale. Les biocarburants sont un atout pour réussir notre transition énergétique ; ils sont un moyen utile pour décarboner les transports, le seul existant à court terme pour les avions. Avec 20 000 emplois directs, ce sont des filières hautement compétitives : la France est ainsi classée au premier rang européen et au cinquième rang mondial pour la production de bioéthanol, au deuxième rang européen et au sixième rang mondial pour celle de biogazole. Enfin, loin d'opposer usages agricole et industriel, les biocarburants concourent à notre indépendance protéique, puisqu'ils permettent la coproduction de drêches et de tourteaux utilisés pour la consommation animale.

l'amendement n° 293 rectifié . Cet amendement vise à donner les moyens d'une relance verte aux territoires. Il prévoit qu'une fraction du produit de la TICPE soit affectée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements,

Dantec, a été voté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2017, puis supprimé par l'Assemblée nationale en seconde lecture. Le Gouvernement repousse le moment de la décision ; les collectivités territoriales, elles, continuent d'avancer sur ces questions. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux : réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre ; réduction de 50 % de la consommation d'énergie finale augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie ; rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017. Mais force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux, votés par une grande majorité des parlementaires, ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l'énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. En France, l'élaboration et la mise en oeuvre des PCAET à l'échelle des à l'échelle des intercommunalités, du volet énergie des Sraddet et des SRCAE à l'échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique. Mais les collectivités territoriales compétentes se sont vu se sont vu transférer de nouvelles compétences, sans aucun transfert de moyens. Or, en l'absence de moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en oeuvre et risquent de rester, en grande partie, à l'état d'intentions. Le présent amendement vise donc à doter les collectivités chargées de l'élaboration et de la mise en oeuvre des PCAET et des Sraddet d'un montant de 10 euros par habitant pour les EPCI et de 5 euros par habitant pour les Sraddet. Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu'en 2018, représentant aujourd'hui 8 milliards d'euros de recettes. Le mouvement des « gilets jaunes » a toutefois marqué un coup d'arrêt à l'augmentation de cette fiscalité. Celle-ci a en effet été, on le sait, vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de la non-affectation des recettes à la transition énergétique.

Bigot. Cet amendement vise à créer une taxe applicable à tous les produits non alimentaires mis sur le marché et ne pouvant pas faire l'objet d'un recyclage. La crise du covid-19 a mis en exergue les limites de notre système économique actuel, tourné vers le consumérisme, la surexploitation de nos ressources naturelles et le manque de prise en compte de notre environnement dans nos politiques publiques. La communauté scientifique s'accorde ainsi sur le fait que l'émergence de pandémies, telles que celle du covid-19, trouve ses origines dans les activités humaines. Il est donc temps d'amorcer un changement radical dans nos modes de production et de consommation. Le présent amendement

qui a bien voulu reprendre une partie de ma proposition de loi concernant la Fondation du patrimoine pour l'inscrire dans ce projet de loi de finances rectificative. Cette proposition de loi avait été votée à l'unanimité au Sénat, puis à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Malheureusement,

aux immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural en dehors du champ d'application géographique défini pour le patrimoine de proximité est susceptible d'engendrer un important effet d'éviction pour ce dernier, en l'absence de définition légale de cette notion. Or ce label a pour objet de conserver ledit patrimoine de proximité, et le champ d'application géographique défini lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale permet, en l'état, de remplir cette mission efficacement à nos yeux. De plus, une extension aux immeubles non visibles, que le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public, nous paraît source d'incohérence avec le régime actuellement applicable et entraînerait un coût supplémentaire pour les finances publiques. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements. Je mets

pour ne pas dire tous, non conformes au droit communautaire. J'ajoute que nous sommes le pays en Europe qui se caractérise par le plus grand nombre de niches de taux de TVA réduits, ce qui nous amène à avoir un taux moyen de TVA

Par cet amendement, nous souhaitons faciliter la vente en vrac en grande surface, exonérer les produits alimentaires et baisser la TVA sur les produits non alimentaires. Nous estimons que cette filière doit être encouragée afin de trouver sa place et se développer. Certes, j'ai bien écouté ce qui vient d'être dit, mais

place un mécanisme qui nous semble juste : augmenter la TVA sur les produits de luxe et la mettre à zéro sur les produits de première nécessité. C'est un débat que nous avons déjà eu dans cet hémicycle.

afin d'abaisser le seuil de rentabilité, comme l'a mentionné d'ailleurs le Président de la République dans son adresse aux professionnels du tourisme, le 25 avril 2020. Il s'agit de redonner des marges de manoeuvre aux professionnels.

lorsqu'il dit qu'il ne croit pas au caractère provisoire d'une diminution du taux de TVA dans le contexte que nous connaissons. De surcroît, il est important pour l'État de conserver des bases de TVA qui soient suffisamment solides pour faire face à ses engagements. Telles sont les raisons pour lesquelles je réitère mon avis défavorable sur la totalité des amendements, à moins qu'ils ne soient retirés.

dernière, en appliquant un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les biens d'occasion reconditionnés ou composés entièrement de matériaux recyclés ou biosourcés.

En matière de baisse de TVA, si la perte de recettes pour l'État est certaine, le bénéfice pour les consommateurs est incertain. Est-ce que vous pensez que la baisse de quelques centimes sera répercutée sur le consommateur ? J'ai le plus grand doute. Je rappelle que le taux de TVA doit viser

Guillaume Gontard, pour présenter l'amendement n° 872. Il s'agit d'un amendement récurrent de notre groupe visant à abaisser le taux de TVA à 5,5 % pour les transports publics réguliers de voyageurs urbains ou interurbains. Nous l'avons proposé en toutes occasions, à chaque loi de finances, dans différentes propositions de loi, sous forme d'amendements, notamment dans la LOM ou encore lors du Pacte ferroviaire.

L'objectif, vous l'aurez compris, est de diminuer le coût du transport public. Cette baisse du taux de TVA serait bénéfique pour l'ensemble des autorités organisatrices, qui, à cause des hausses précédentes, ont perdu près de 220 millions d'euros. Elles pourraient décider d'en faire profiter les usagers, comme le propose la Convention citoyenne pour le climat, ou d'utiliser les sommes économisées pour régénérer le matériel ou améliorer l'offre. Cet amendement avait même obtenu l'adhésion de la majorité du Sénat lors de la discussion de l'une de nos propositions de loi. Il s'agit également, d'une sollicitation de l'Association des régions de France. Une telle mesure correspond aussi à l'une des préconisations du rapport récent sur la gratuité des transports. Son adoption permettrait enfin d'envoyer un signal clair en direction de la Convention citoyenne

amendement, comme le précédent, vise à considérer le transport public comme un produit de première nécessité, compte tenu du rôle social essentiel qui est le sien et de sa contribution à la réalisation d'objectifs de transition écologique. En janvier, l'Allemagne a adopté une mesure similaire

de rendre plus attractif le train, dont on sait qu'il est peu émetteur de gaz à effet de serre et générateur d'externalités positives. Le train constitue l'un des moyens essentiels pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l'horizon de 2050. Par ailleurs, une politique tarifaire rendant plus accessible le train favorise la mobilité pour tous et constitue un facteur de lutte contre les exclusions sociales. Il est donc primordial que le train soit désormais considéré comme un service de première nécessité. Une telle politique permet aussi, dans l'absolu, de favoriser le report modal vers le train. Pour toutes ces raisons, nous proposons de réduire le taux de TVA imputé sur le prix des billets de transport de personnes de 10 % à 5,5 %.

Filleul. Nous proposons d'abaisser le taux de TVA imputé sur le transport fluvial de marchandises et de voyageurs à 5,5 % pour engager une diminution des prix favorisant ce mode de transport. Un des objectifs fixés par la Convention citoyenne pour le climat réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de longues distances en permettant un report modal vers le ferroviaire ou le fluvial. La crise sanitaire a prouvé, s'il le fallait, que notre écosystème est très fragilisé par nos modes de production, de consommation et de déplacement. Il y a urgence à mettre en oeuvre la transition écologique. Le transport, avec 33 % des émissions, est le secteur le plus concerné par cette nécessaire transition. Pour respecter nos engagements et atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l'horizon de 2050, il est urgent de de développer les mobilités durables. Le transport fluvial en fait partie, mais il est souvent, malheureusement, le grand oublié des politiques publiques. La France est le pays européen avec le plus grand nombre de canaux navigables, mais ceux-ci sont paradoxalement les moins fréquentés, alors que nos routes saturent.